des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2024 rapport n° 84, avis n° 80). Mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s’effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle ci fonctionne correctement en l’insérant dans votre terminal de vote. Vous pourrez vous rapprocher des huissiers pour toute difficulté. Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.

à la santé des femmes et une modification du financement des hôpitaux dont nous approuvons le principe et attendons les modalités. Toutefois, ces mesures ne peuvent faire oublier le cadre général restrictif, la procrastination politique sur la dépendance et l’inexistence de politiques affirmées sur la famille et sur les accidents du travail et maladies professionnelles (AT MP). Ces deux derniers sujets souffrent du désintérêt ancien pour la prévention. En définitive, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) est décevant, car il n’impulse aucun des changements profonds indispensables au maintien d’un système solidaire.

qui impose d’affronter avec volontarisme les consommations de tabac et d’alcool, les facteurs environnementaux, la qualité de notre alimentation et l’activité physique. il ne contient aucune mesure de nature à freiner la financiarisation du système de santé, qui transforme les cotisations des assurés sociaux en revenus pour actionnaires. Comment, dans de telles conditions, prétendre agir sur la pertinence des soins ? loi laisse les pénuries multiples se répandre. Vous l’aurez compris, nous estimons, madame, monsieur les ministres, que le budget que vous nous présentez est une impasse. La crise sanitaire qui a frappé en 2020 est derrière nous, mais les enseignements ne sont pas tirés. Alors qu’il faudrait réunir un large accord politique pour rénover en profondeur notre protection sociale et notre système de santé, la faiblesse de votre base en la matière empêche le Parlement de remplir pleinement son rôle.

J’évoquerai avec vous mes regrets, qui sont à la hauteur du devoir qui nous incombe. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est un aveu d’impuissance sur le plan budgétaire.

Déjà plus important que l’an dernier, le déficit devrait se creuser au cours des prochaines années pour atteindre plus de 17 milliards d’euros en 2026 et en 2027. Pour cette raison, le groupe Les Républicains rejoint l’analyse de la commission des affaires sociales du Sénat sur la trajectoire financière de ce PLFSS, dont nous déplorons l’insincérité et l’incohérence.

ni de détailler les économies prévues à hauteur de 3,5 milliards d’euros. En témoigne explicitement la hausse des franchises et de la participation forfaitaire, au traitement malheureusement trop caricatural. Si le soutien à la vaccination contre le papillomavirus humain est le bienvenu, il constitue la seule mesure de prévention tandis que la prescription d’antibiotiques par les pharmaciens contre les angines et contre les cystites est la seule en matière d’amélioration de l’accès aux soins. Mes chers, collègues, la prévention et l’amélioration de l’accès aux soins ne peuvent en rester là

Je vous parlais de regrets. En voilà un autre : la profonde, voire inquiétante, impréparation du Gouvernement sur ce texte. Puisque nous avons jugé que la réforme du financement de l’hôpital était trop précipitée, nous avons reporté son entrée en vigueur au 1 janvier 2028, après trois années d’expérimentation, pour ne pas mettre en danger les hôpitaux. Nous ne pouvons que regretter la méthode du Gouvernement, qui, sans étude d’impact ni financements complémentaires, entend poursuivre une ambition dénuée de prudence. Mes chers collègues, refusons de jouer avec l’hôpital pour des effets d’annonce

allée de pair avec l’impréparation, se retrouve par ailleurs dans l’abandon à mi chemin de l’article 39. La suppression pure et simple de ce dernier est la brillante démonstration de mesures mal anticipées, concoctées à la hâte. Un temps de concertation supplémentaire est souhaitable, voire nécessaire, avant d’adopter des modifications aussi substantielles sur le régime de la rente AT MP. La branche famille est la grande oubliée de ce projet Grâce aux modifications du Sénat, elle se voit transférer 2 milliards d’euros issus de la branche maladie. Ce montant répond au précédent transfert, depuis l’assurance maladie maternité, de la charge du congé de maternité postnatal. Cette mesure, qui répondait à une logique comptable, masque un manque d’ambition en faveur de la politique familiale : ce congé, pas plus que la grossesse, n’est un mode de garde ; par contre, il relève bien de la santé ! Tant qu’il n’y aura pas de budget pour soutenir les familles, il n’y aura pas de véritable politique nataliste dont le pays a pourtant que représentaient certaines mesures. En voici une, proposée par le groupe Les Républicains : la possibilité, pour les orphelins dont les parents sont affiliés au régime des artisans, des commerçants et des professions libérales, de bénéficier d’une pension de réversion. Si cette mesure de justice sociale visait déjà les fonctionnaires et les salariés du privé depuis l’année dernière, notre groupe a élargi les critères d’éligibilité à la pension de réversion des orphelins en situation de handicap éloignés de l’emploi.

la prestation de compensation du handicap (PCH) et pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Nous avons adopté la proposition du Gouvernement de verser aux départements un complément au concours APA de 150 millions d’euros et de transformer en expérimentation la fusion des sections soins et dépendance pour le financement des Nous regrettons, hélas !, que ces montants soient bien en deçà des besoins financiers des départements, surtout si le Gouvernement s’en tient à sa proposition de 150 millions d’euros. Nous attendons toujours de pied ferme une réforme sur le financement du secteur de la dépendance et du handicap. Nous avons aussi renforcé les droits des élus locaux en matière de retraite. Depuis le 1 septembre 2023, l’ensemble des élus peuvent cotiser au régime général sur ces indemnités après une simple demande auprès de leur collectivité. Nous avons désormais intégré à ce champ les délégués des collectivités territoriales membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin de parachever l’avancée en matière de droits à la retraite. Nous nous réjouissons également de la suppression de la disposition prévoyant une contribution de l’Agirc Arrco au système de retraite. L’État n’a pas à ponctionner les caisses de ces complémentaires, constituées de l’excédent obtenu par les efforts des salariés. Si l’État souhaite financer de nouvelles dépenses, qu’il fasse des économies.

C’est pourquoi nous voulons rendre obligatoire d’ici à trois ans le contrôle biométrique des retraités résidant à l’étranger et intégrer des agents des conseils départementaux aux échanges d’informations entre agents de l’État et organismes de protection sociale. Nous devons continuer sur cette voie et faire de la lutte contre la fraude à l’assurance maladie un cheval de bataille. Parce que les Français méritent que nous parlions de santé, de prévention, de politique familiale et du bien vieillir, parce que nos aînés attendent que nous trouvions des solutions pour la prise en charge du grand âge et de la dépendance, parce que l’ensemble des professionnels méritent que nous discutions du déficit budgétaire des établissements de santé et des établissements médico sociaux, parce que les familles méritent que nous nous orientions vers une politique nataliste et vers une meilleure conciliation

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, à la lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons l’impression d’être, comme l’arche de Bercy, noyés dans la Seine et de continuer la brasse coulée de ces dernières années. La balance sociale est toujours aussi déséquilibrée. Les dépenses, qui atteignent 255 milliards d’euros, sont en hausse de 3,2 % par rapport à 2023 ; le déficit, quant à lui, est amené à se creuser à 17,5 milliards d’euros d’ici à 2027, selon vos prévisions les plus optimistes. Alors qu’environ 60 % des Français auraient déjà renoncé à se soigner, en raison soit de délais d’attente soit du coût de la consultation, vous vous apprêtez à ajouter un impôt sur la santé en augmentant la franchise à la charge des patients sur les boîtes de médicaments et sur les consultations. Dans la ruralité comme dans les métropoles, les maternités et les services d’urgences ferment épisodiquement, pour ne pas sombrer, ou définitivement. La France des hôpitaux recule. Les déserts médicaux progressent. Malgré cela, vous imposez une austérité de 600 millions d’euros aux Pour dégrossir la bête, vous choisissez de retirer le squelette au lieu de réduire les graisses. Pendant que le soin et l’accueil de la vie reculent, l’idéologie progresse. Le système de sécurité sociale, auquel nous cotisons tous très largement, rembourse les transitions de genre et les détransitions qui s’ensuivent. Oh ! là là ! L’État finance également des « salles de shoot », qui se trouveront bientôt dans nos rues à Marseille, alors qu’à l’approche de l’hiver certains médicaments de première nécessité, comme l’amoxicilline, manquent dans de nombreuses pharmacies. Nous sommes très loin des inspirations du catholicisme social à l’origine de notre modèle de protection sociale. L’idéologie a pris le pas sur la solidarité J’en veux encore pour preuve le fait que, le 1 octobre dernier, la prise en charge des soins dentaires par l’assurance maladie est passée de 70 % à 60 % quand, dans le même temps, vous proposez la gratuité des préservatifs et des protections hygiéniques pour les moins de 26 ans. Le socialisme vous aveugle ! Vous êtes les ministres Vous êtes les ministres chargés de financer la santé des Français, pas leur sexualité ! Il faut revenir au régalien et cesser de régaler ! Le pire est encore à venir avec le projet de loi sur l’euthanasie, visant à éliminer les coûteux pensionnaires du système de sécurité sociale là où vous vous trouvez incapables de contribuer au bien vieillir. Enfin, alors que les départements peinent à soutenir les structures d’aide à domicile et les Ehpad, vous avez déclaré, monsieur le ministre, que la Cour des comptes ne pouvait connaître le détail du nombre de cartes Vitale en circulation dans notre pays. Dans quel genre de régime vivons nous ? En l’absence de transparence et de contrôle, nous sommes obligés de croire que les chiffrages actuels sont minimalistes. Pourtant, ils annoncent 75 millions d’assurés sociaux en France pour 67 millions d’habitants, soit 8,2 millions d’assurés sociaux en trop dans le système ! La fraude sociale est La fraude sociale est la seule industrie qui se développe encore dans notre pays. Elle est une gigantesque injustice nationale et sanitaire. Il faut conclure ! Sans aucune évolution dans ce domaine et malgré les avancées du Sénat, je me refuserai à donner mon aval à votre texte.

cette année encore, l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale a été l’occasion de débats importants sur l’orientation budgétaire que nous souhaitons donner à notre pays en la matière.

Cet abîme de milliards au dessus duquel nous nous penchons doit nous alerter sans pour autant nous conduire à l’immobilisme en matière de protection sociale. La peur de continuer à creuser le déficit doit toutefois guider nos choix, les bons, ceux ceux qui permettront aux Français de continuer de bénéficier de la sécurité sociale dans les meilleures conditions, sans risquer de remettre en question l’existence même de ce qui fait la force de notre République. C’est exactement le choix qu’avait fait le Sénat, en mars dernier, en adoptant le recul de l’âge de départ à la retraite tout en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité ou encore de la maternité. Cette réforme n’empêchera pas à court terme la branche retraite de creuser son déficit. Elle illustre la capacité du Sénat à prendre ses responsabilités et les mesures qui s’imposent, aussi impopulaires soient elles, pour sauvegarder notre système de retraite. Premièrement, ce texte contient des avancées très concrètes pour nos concitoyens grâce à la prise en charge des préservatifs et des protections féminines réutilisables pour les jeunes, la possibilité pour les pharmaciens de délivrer, dans un cadre précis, certains médicaments de première urgence sans prescription médicale ou encore à la simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire. Ces mesures représentent des apports dont beaucoup de Français pourront bénéficier et il est bon de constater qu’un consensus peut exister au moins sur ces sujets. comme tous ici, certainement, nous partageons l’idée selon laquelle la clé de voûte de tout système de santé doit être la prévention. Nous nous réjouissons des précisions que le texte apporte concernant les rendez vous de prévention aux âges clés de la vie et de la proposition de vaccination dès le collège contre le contre le papillomavirus humain, surtout au regard de l’efficacité du vaccin lorsqu’il est administré avant le début de la vie sexuelle. Sur le terrain de la prévention, nous avons suivi avec intérêt les débats autour d’une plus forte taxation des boissons et des produits sucrés. sucrés. La question mérite d’être posée, même si nous ne pensons pas nécessairement que l’augmentation des taxes soit la meilleure réponse à apporter à un problème de santé publique.

ce texte prévoit le renforcement du contrôle des arrêts de travail. Leurs répercussions sur les comptes de la branche maladie sont une réalité. Que l’augmentation de leur coût soit due à l’évolution de leur nombre ou à celle du montant des indemnités journalières, il faut prévoir un meilleur encadrement pour éviter les abus

le texte contient des outils de lutte contre la fraude aux cotisations sociales. À ce titre, nous regrettons que l’article 6, qui concernait les microentrepreneurs de plateformes numériques, ait été supprimé. Nous regrettons également que le texte ne soit pas à la hauteur du défi de la dépendance. Sur ce point, la réalité dépasse nettement les ambitions. Le nombre de seniors de plus de 85 ans doublera d’ici à 2040. L’ensemble des emplois promis auprès de nos aînés doivent être créés dès maintenant et non pas lors du prochain quinquennat. Nous regrettons, en outre, que le texte soit quelque peu lacunaire sur le développement des soins palliatifs.

Si ce montant nous semblait insuffisant pour les hôpitaux comme pour le secteur médico social, nous ne partageons pas les raisons invoquées ayant conduit à la suppression des articles en question vendredi dernier. Le groupe Les Indépendants – République et

Un pays qui s’endette pour financer sa protection sociale, un pays qui reporte le financement de sa protection sociale sur les générations futures est un pays qui va mal, très mal. Or ce pays, c’est la France ! Madame, monsieur les ministres, je crains que l’histoire ne juge sévèrement cette période d’endettement public. Ce PLFSS ne prend pas en compte le changement de monde, la fin de l’argent pas cher et la hausse des taux d’intérêt.

Mais tout est dans. N’est ce pas, monsieur le ministre ? Alors, quelles solutions ? À gauche, j’ai écouté Bernard Jomier. C’est toujours la même réponse : l’augmentation des prélèvements, souvent en préconisant la suppression des exonérations de charges patronales et salariales.

Si ces remarques peuvent s’appliquer à toutes les branches, elles concernent en priorité la branche maladie. Il faut revoir notre organisation pour la médecine de ville, ainsi que notre organisation et notre management du système hospitalier.

l’occasion d’une recentralisation par le transfert de la tutelle des Ehpad sur les agences régionales de santé (ARS). Pour nous, le département doit encore renforcer sa place d’organisateur de l’action sociale dans la totalité de ses composantes. Pour la branche autonomie, il y a urgence à aborder courageusement une loi autonomie pour le grand âge et le handicap sur le plan des moyens, mais aussi de la gouvernance.

et des carrières hachées. C’est une réalité. Merci René Paul Savary ! Enfin, la branche famille est la grande oubliée ! Rien ou presque rien sur le tiers payant du complément de mode de garde, sur le congé parental, sur l’universalité des allocations familiales ou sur le service public de la petite enfance. Cette pauvreté de la politique familiale est une nouvelle illustration que ce gouvernement n’est pas suffisamment tourné vers l’avenir, alors même que notre natalité chute de 850 000 naissances à 700 000 naissances. Mes chers collègues, le PLFSS demeure un texte financier. Son équilibre, ou plutôt son absence d’équilibre résulte de choix ou de non choix

L’ensemble des travées, ou presque, ont répondu « non ». L’Ondam a t il été piloté depuis la crise sanitaire ? Le Gouvernement a répondu « non L’Ondam tel qu’il est présenté au Parlement est il un outil démocratiquement satisfaisant ? Encore « non » ! Notre groupe a rejeté l’Ondam. Toutefois, contrairement à la majorité sénatoriale, il ne s’agissait pas de sanctionner une dérive de l’Ondam ou de condamner des dépenses excessives d’assurance maladie. Que d’hypocrisies lors de notre débat ! Alors que le déficit de la sécurité sociale s’aggrave au fil des années et atteint 8,8 milliards d’euros en 2023, la majorité sénatoriale et le Gouvernement ont rejeté nos propositions de nouvelles recettes. Notre amendement visant à créer une cotisation sur les superprofits aurait rapporté à lui seul 10 milliards d’euros de recettes pour la sécurité sociale et aurait rétabli, sans aucune autre taxe, une justice sociale nécessaire. Ainsi, faute de perspectives avons nous rejeté l’Ondam, en l’absence d’une trajectoire claire de financement permettant de garantir la sécurité sociale, face à une voie illusoire dans ses moyens et sans issue dans sa réalité. Soyons précis. Quel défi fallait il relever pour sauver notre sécurité sociale et répondre aux enjeux d’avenir ? Je vous parle là d’une réalité : urgences hospitalières engorgées, difficultés pour trouver un médecin généraliste en secteur 1, possibilité moindre de bénéficier d’une retraite avant de mourir, accès aux soins réduit lorsqu’on n’est pas français, inégalité devant l’achat d’un fauteuil roulant. Je vous parle simplement de notre contrat social de solidarité, de fraternité et d’égalité. Je le répète, je sais que, dans cet hémicycle, y compris sur les bancs du Gouvernement, nous sommes nombreuses et nombreux à partager l’idéal de cette conquête sociale, à nous battre pour que les plus précaires aient accès aux droits fondamentaux, à souhaiter que la sécurité sociale soit garantie. Or ce texte n’apporte aucune solution à la désertification médicale, aux problématiques d’accès aux soins,

notre pays, des milliers de professionnels de santé. En un mot, face à l’urgence écologique, sociale, et économique, il eût fallu un virage majeur pour préserver la sécurité sociale et protéger les plus précaires. Or ce texte ne l’amorce pas. ressemble plus à un bricolé qu’à un plan de financement. Soyons clairvoyants ! Le Gouvernement engagera sa responsabilité devant l’Assemblée nationale pour faire adopter le texte budgétaire qu’il souhaite. Pauvre démocratie ! Je compte sur vous, monsieur le ministre, madame la ministre, pour protéger, pour le moins, les mesures utiles que nous avons intégrées à ce projet de loi et que nous pouvons partager, quels que soient nos désaccords, notamment en termes de prévention. l’intensification de l’information et de la sensibilisation dans les établissements scolaires pour que la campagne vaccinale contre le virus du papillome humain soit un succès, à l’amélioration de la continuité de la prise en charge des frais de santé des Françaises et des Français de l’étranger qui viennent se réinstaller en France, la création d’une taxe sur les publicités pour les jeux d’argent et de hasard, à la suppression de la ponction dans les caisses d’assurance chômage ou encore au maintien de la contribution tarifaire d’acheminement vers la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des pensions de retraite. certains enjeux majeurs de la santé et de la protection sociale n’ont pas pu être correctement discutés la semaine dernière et ont été finalement balayés. Nous ne pouvons pas faire l’économie de la santé environnementale, de la démocratie sanitaire, de la réduction des risques, de la santé communautaire et de la lutte contre les addictions. Autant de sujets dont le texte ne s’empare pas

Vous l’aurez compris, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires considère ce texte insuffisant pour répondre aux enjeux contemporains de la santé et de la protection sociale. Malgré quelques mesures de prévention et le début d’une autre tarification hospitalière, ce projet de loi propose un.

Pour la santé et le social, comme pour le climat, il n’y a pas de ! Il y a un naufrage annoncé, et nous voguons à bord d’un Titanic que nous croyons insubmersible, mais qui, sans prise de conscience rapide, coulera assurément. assurément. Préparons nous ! Il y a urgence pour garantir notre sécurité sociale et environnementale. Notre groupe votera donc contre ce texte. La

nous avons achevé l’examen du budget de la sécurité sociale pour 2024. Durant cinq jours et quatre nuits, nous avons examiné 830 amendements portant sur un budget de 640 milliards d’euros. Quel bilan tirons nous de ces débats ? La copie du Gouvernement, adoptée à l’Assemblée nationale avec un passage par le 49.3, était très médiocre et, surtout, largement insuffisante. Nous l’avons dénoncée au cours de nos interventions. Le budget de la santé est largement insuffisant pour répondre aux difficultés rencontrées dans les hôpitaux, aux difficultés liées aux pénuries de médicaments, aux difficultés pour avoir un rendez vous avec un médecin. Les budgets des branches famille et accidents du travail maladies professionnelles sont également sous dotés et dénués de vision politique ambitieuse, ce qui est très regrettable. Le budget pour 2024 de la branche autonomie est aux antipodes des besoins rencontrés par le secteur médico social et aux antipodes des futurs besoins engendrés par le vieillissement de la population. Enfin, le budget de l’assurance vieillesse démontre l’inefficacité de la contre réforme des retraites, qui devait permettre le retour à l’équilibre et qui aggravera finalement le déficit de 12 milliards d’euros en 2027. Le Gouvernement a équilibré le budget de la sécurité sociale pour 2024 par des mesures d’économies réalisées sur le dos des assurés sociaux, en renforçant par exemple les contrôles des arrêts maladie ou en déremboursant les soins dentaires. Que devons nous retenir des modifications apportées par la majorité sénatoriale ? Tout au long de l’examen de ce PLFSS, le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont, d’une même voix, rejeté par dogmatisme tous nos amendements prévoyant de nouvelles recettes. Nous avons proposé pour notre part de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations patronales, ce qui rapporterait 8 milliards d’euros. Nous avons proposé de mettre à contribution les bénéfices records réalisés par les entreprises, en créant une contribution des revenus financiers, sociale généralisée (CSG) sur les produits financiers et en créant une contribution de solidarité des actionnaires, ce qui rapporterait près de 40 milliards d’euros. Nous avons proposé d’instituer une contribution sociale exceptionnelle sur les sociétés réalisant des superprofits, ce qui rapporterait 10 milliards d’euros. Nous avons proposé d’instituer l’égalité salariale femmes hommes, ce qui rapporterait 5 milliards d’euros. nous avons proposé de supprimer les exonérations de cotisations sociales, ce qui rapporterait 87,9 milliards d’euros. Vous avez refusé 150 milliards d’euros de recettes supplémentaires, pour des raisons dogmatiques de défense des entreprises et des plus aisés.

Comment ne pas être en colère face à l’incapacité du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de tirer les conséquences de l’échec des politiques de réduction des dépenses ? Si les hôpitaux publics subissent une désertion en masse des professionnels de santé, c’est en raison de la dégradation de leurs conditions de travail. Des décennies de coupes budgétaires ont imposé un travail de plus en plus pénible dans les hôpitaux. Ceux ci sont devenus des organisations maltraitantes qui usent les personnels et dégradent la qualité des soins. des secteurs de la santé et du médico social sont pourtant profondément attachés au service public et à la qualité de la prise en charge des patientes et des patients. Notre modèle de sécurité sociale est dangereusement remis en cause par les exonérations de cotisations patronales. dénonce pression fiscale et montant des cotisations sociales. Pourtant, les exonérations patronales n’ont jamais été aussi importantes ! La réduction des cotisations patronales, actée encore récemment

Après le vote du Sénat, le Gouvernement pourra dégainer une dernière fois le 49.3 à l’Assemblée nationale lors de l’examen en nouvelle lecture du PLFSS 2024. Cela ouvrira le bal des textes financiers sur lesquels les députés seront privés de vote. En conclusion, ce PLFSS 2024 est un rendez vous manqué pour un financement à la hauteur des besoins sociaux, mais aussi un rendez vous manqué pour reprendre la main sur la maîtrise publique de la production de médicaments. Lors de nos débats, le président de la commission des affaires sociales a souligné à plusieurs reprises son souhait que la commission « se saisisse » de certains dossiers. Sachez que nous sommes volontaires pour y participer. Pour l’ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, qui ont défendu un autre projet que le vôtre

642 milliards d’euros de dépenses et 631 milliards d’euros de recettes : voilà l’essentiel de ce que nous nous apprêtons à voter. C’est un budget colossal, marqué par un déficit tout aussi colossal de plus de 10 milliards d’euros l’an prochain. Alors que nous approchions l’équilibre avant le covid 19 et que nous espérions une amélioration avec la fin de la crise sanitaire et la réforme des retraites, les prévisions pour les années à venir ne sont pas très optimistes. L’annexe A de ce projet de loi prédit un déficit des branches maladie et vieillesse plus élevé en 2027 qu’en 2024, alors même que les prévisions de croissance seraient surestimées, d’après l’analyse du Haut Conseil des finances publiques. Une telle trajectoire a été rejetée par la grande majorité des membres Pour notre groupe, ce rejet traduit notre inquiétude sur la soutenabilité de notre système de santé, notre inquiétude pour les générations futures, à qui nous transmettons cette dette, et notre inquiétude relative à une financiarisation de la santé.

et augmenter les recettes sans porter atteinte à la compétitivité de nos entreprises ni dégrader le pouvoir d’achat de nos concitoyens, le champ d’action est particulièrement étroit. À l’horizon 2050, la population française comptera près de 20 millions de personnes âgées, dont 4 millions seront en perte d’autonomie. À cela s’ajoutent l’explosion des maladies chroniques et l’arrivée de nouvelles thérapeutiques innovantes, plus coûteuses. C’est une évidence : nous aurons besoin de plus de soignants, à qui nous devrons proposer de bonnes conditions de travail. Il n’est donc pas difficile de comprendre que certaines dépenses de santé continueront de croître. Pour autant, nous ne pouvons pas laisser la situation se dégrader encore sous nos yeux. Nous sommes ainsi convaincus qu’un travail de fond et de long terme doit être mené. Nous devons examiner courageusement et sans tabou la pertinence des soins. Le coût de la gestion administrative de notre système de santé est pointé du doigt par la Cour des comptes. Selon cette dernière, si le système français a l’avantage de garantir un « reste à charge particulièrement faible », il est « particulièrement coûteux en frais de gestion Elle préconise aussi de faire en sorte que les financements de la sécurité sociale et des mutuelles, dont les frais de gestion augmentent, ne se superposent plus, ce qui est souvent le cas à l’heure actuelle. La suradministration représente 5,6 % des dépenses totales de santé, notamment du fait de la trop grande centralisation de notre système. Nous devons aller plus loin dans la décentralisation, faire confiance aux territoires et acteurs de terrain, comme d’autres pays en Europe s’y sont employés. En attendant, des pistes de réduction des dépenses existent. Outre les mesures de lutte contre la fraude, bien enrichies par le Sénat, l’accent doit surtout être mis sur la prévention et l’éducation à la santé. Nous soutenons toutes les mesures qui vont dans ce sens. Sur la vaccination contre le papillomavirus, la campagne nationale menée dans les collèges est une excellente initiative, de même que sa généralisation dans ce PLFSS. En effet, le papillomavirus est à l’origine de 6 400 nouveaux cas par an. C’est un véritable enjeu de santé publique. Vaccination et dépistage peuvent ouvrir la perspective d’une éradication du cancer du col de l’utérus. Compte tenu de la forte désinformation concernant ce vaccin, de la peur agitée sur des risques supposés, mais jamais démontrés, nous insistons sur l’importance de renforcer l’information des jeunes et de leur famille en amont des campagnes de vaccination. C’est l’objet d’un amendement qui a été adopté. À titre personnel, mon incompréhension demeure quant au rejet de toute taxe supplémentaire sur l’alcool, alors que la méthode a montré son efficacité pour le tabac et que l’on connaît parfaitement les risques majeurs que la consommation d’alcool fait peser sur la santé. À l’origine de 41 000 décès par an en France, deuxième cause de mortalité évitable, l’alcool coûte 102 milliards d’euros par an à la société. Plus de recettes pour la prévention, moins de dépenses pour des maladies graves qui seront évitées : tels sont les enjeux de la taxe comportementale, qui ne doit pas être opposée

Toujours en matière de prévention, nous nous félicitons de voir enfin un premier pas fait en faveur du remboursement de l’activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer. C’est un sujet que je défends de longue date, et je suis satisfaite de voir l’amendement de notre groupe adopté, avec le soutien du Gouvernement et de la commission. de la commission. Pour les autres mesures visant à réduire les dépenses, je soutiens à titre personnel certaines dispositions du texte issu de l’Assemblée : l’application sans délai de la réforme de la tarification à l’activité (T2A), l’interdiction de prescrire des arrêts de travail de plus de trois jours en téléconsultation, l’incitation aux transports sanitaires partagés ou encore la délivrance de médicaments à l’unité, en cas de rupture d’approvisionnement. Ce sont des mesures de sobriété et de bon sens, dont certaines, et je le regrette, ont été supprimées. Nous nous réjouissons de l’adoption de certains amendements que nous avons défendus. Il s’agissait d’amendements de justice, de cohérence et de simplification, visant

la suppression du coefficient de minoration pour les établissements privés à but non lucratif. Il pénalise injustement les centres de lutte contre le cancer et des hôpitaux, qui, sur de nombreux territoires, dont le mien, assurent seuls les missions de service public auprès de la population. J’aimerais également vous parler de mon département, qui se trouve aux frontières de la Belgique et du Luxembourg. Nous subissons une double peine : outre la situation nationale de pénurie de soignants, la concurrence frontalière fragilise grandement nos hôpitaux et nos soins de premier recours. Nos professionnels de santé sont « aspirés » – le mot n’est pas beau, mais il reflète bien la réalité – par le Luxembourg, où les salaires sont jusqu’à trois fois plus élevés. J’ai proposé par amendement la prise en compte de la concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique. Si cet amendement a été rejeté, le ministre a semblé ouvert à d’autres pistes.

Ce texte s’inscrit dans un contexte difficile – nous l’avons dit – pour notre système de santé, fragilisé par une inflation forte et une augmentation de ses coûts de fonctionnement. L’objectif du texte était clair : soutenir les établissements de santé les plus fragiles, permettre au personnel soignant de gagner dignement sa vie sans que les avancées du Ségur soient effacées, moderniser et mieux prendre en charge les patients dans notre pays. Un objectif, et un horizon la maîtrise des dépenses et du déficit, et la recherche d’économies, quand c’est possible, dans les différentes branches, notamment pour les soins de ville. Sont prévus également le soutien aux plus précaires avec la simplification de l’attribution de la complémentaire santé solidaire, réforme du financement des hôpitaux, l’intensification de la lutte contre la fraude sociale, le renforcement des compétences des pharmaciens et la lutte contre les pénuries de médicaments… Les avancées contenues dans ce texte sont nombreuses. Deux orientations, en particulier, sont à souligner : le soutien à l’autonomie et le renforcement de la prévention. Sur le soutien à l’autonomie, 39,9 milliards d’euros seront engagés en 2024 pour renforcer l’attractivité des métiers, adapter l’offre médico sociale aux besoins démographiques et améliorer la qualité des accompagnements. Soulignons notamment la mise en place, désormais sous la forme d’une expérimentation, d’une fusion des sections « soins » et « dépendances » dans certains départements, en vue de la création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile. le renforcement de la prévention, 150 millions d’euros supplémentaires sont destinés à la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus ou la prise en charge intégrale des protections périodiques réutilisables et des préservatifs pour les moins de 26 ans. Je tiens par ailleurs à saluer, madame la ministre, l’adoption d’un amendement du Gouvernement permettant la prise en charge du sport sur ordonnance. C’est un signal très positif, qui s’inscrit pleinement dans la grande cause nationale souhaitée par le Président de la République. C’est une mesure que vous savez attendue, tout particulièrement dans les territoires ultramarins. Au cours des débats, notre groupe a formulé un certain nombre de propositions. Nous nous réjouissons de l’adoption de plusieurs d’entre elles. Je pense aux amendements de notre collègue Xavier Iacovelli, qui ont permis d’alourdir la taxation des produits les plus sucrés, afin de ralentir la progression de l’obésité et du diabète et d’inciter les industriels à proposer des produits plus sains. Je pense également à l’amendement permettant à un orphelin handicapé de bénéficier, sans condition d’âge, d’une pension de réversion à la suite du décès d’un ou de ses deux parents. d’un amendement de notre collègue Nadège Havet permettra de poursuivre les efforts engagés en faveur d’une mobilité plus sobre et décarbonée, en facilitant le remboursement des frais de location de vélos par l’employeur.

Mes chers collègues, ces avancées sociales et sanitaires auraient dû conduire notre groupe à voter en faveur de ce projet de loi. Pourtant, nous ne le voterons pas.

lui reprochant tout à la fois de ne pas prévoir ce qu’il ne peut pas prévoir et d’être insuffisamment maîtrisé quand il se révèle chaque année insuffisant. Dans cette même logique, vous avez rejeté la trajectoire des comptes de la sécurité sociale pour les prochaines années,

Nous ne sommes pas non plus convaincus par le report à 2028 de la réforme du financement des établissements de santé et, avec elle, de la T2A. Cette réforme est attendue ; elle est prête. Ayons le courage de la mener. Un mot enfin sur la révision des coefficients géographiques appliqués aux établissements de santé situés dans les territoires ultramarins, et tout particulièrement en Guadeloupe

effacer toutes les craintes. Les professionnels de santé appellent en effet à la création de missions d’intérêt général propres aux outre mer, afin de prendre en compte les défis structurels auxquels ces territoires font face. Je pense notamment à l’accessibilité des établissements ou à la prévalence de certaines maladies chroniques. Au cours de ces cinq jours de débats, c’est au fond la question lancinante de la refonte structurelle du financement de la sécurité sociale qui s’est imposée. Le Gouvernement doit l’entendre. Le Sénat doit s’en emparer.

fourni sur ce texte. Il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l’ensemble du projet de loi, modifié, de financement de la sécurité sociale pour 2024.

quel rôle et quels moyens pour les collectivités locales ? Quel accompagnement du citoyen ? » Dans le

Merci

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la perspective du Congrès des maires, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a souhaité proposer ce débat de contrôle pour interroger le Gouvernement sur les modalités d’accompagnement et de concertation dont s’assortit, pour les collectivités locales, le volet planification de la transition écologique. Les feux hors normes de 2022, les sécheresses qui se sont prolongées jusqu’à l’automne et les inondations que connaît aujourd’hui le nord de la France nous rappellent de façon vive que la transition écologique, au delà des discours, nécessite d’être mise en œuvre selon une fondée sur une planification décentralisée et comprise par tous. Les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes et leurs groupements, les départements et les régions sont donc incontournables. Malheureusement, la présentation par le Président de la République, le 25 septembre dernier, de sa feuille de route écologique n’a pas clarifié les modalités de cette mise en œuvre nécessaire à l’échelle territoriale.

Cette feuille de route, loin de constituer un nouveau départ, est une redite de ce que nous demandions depuis plusieurs années : par exemple, l’annonce de la sortie du charbon, censément entérinée depuis 2022, ou encore la mise en place de RER métropolitains, renommés, grâce à l’action du Parlement, sous le

Les défis sont pourtant immenses : il faut définir le rôle et les compétences des collectivités locales, accompagner le citoyen, faire de la pédagogie lorsque cela est nécessaire et ne pas laisser derrière nous les populations les plus fragiles. créer un récit et embarquer tous nos concitoyens dans l’aventure de la transition écologique, qui est, je le crois, porteuse d’espérance. Une fois interrogée la vision, regardons maintenant du côté des moyens et des outils apportés par l’État. Là encore, nous restons sur notre faim. Les dispositifs présentés manquent cruellement d’une colonne vertébrale territorialisée. La logique d’appels à projets revient à arroser des territoires, sans concertation, sans définition d’une bonne manière d’agir, sans cartographie des besoins.

J’étais ce week end avec l’association des maires ruraux de Gironde pour faire le point. De nombreuses communes se trouvent en grande difficulté pour répondre aux injonctions de l’État, car, estiment elles, elles n’ont eu ni l’ingénierie ni l’accompagnement nécessaires. Or les délais sont très courts. C’est pourquoi il faut créer un cadre de dialogue avec l’État sur la base d’un projet de territoire partagé avec les différents acteurs publics et privés. Ainsi seulement se donnera t on les moyens de faire converger nos projets, les orientations de l’État et les sources de financement. Médiatisées lors du Congrès des régions de France, les COP régionales ont fait leur apparition dans le paysage, un peu à la façon d’un nouveau numéro vert, avec la lourde tâche de « faire converger travaux nationaux et remontées des territoires », pour reprendre les mots de la Première ministre. Ainsi, il serait demandé aux conseils régionaux d’organiser, avec l’État, des COP dans un temps record et de mettre en place un plan d’action avant l’été prochain. Une telle annonce est tout de même surprenante dans la mesure où la plupart des collectivités ou, du moins, un grand nombre d’entre elles n’ont pas attendu le Gouvernement pour se lancer dans une logique de planification.

Comment ne pas imaginer que derrière ce calendrier intenable se cache la volonté du Gouvernement de se désengager d’une partie de la mise en œuvre de la planification écologique en renvoyant aux régions la responsabilité de proposer leur propre feuille de route ?

des blocs infrarégionaux des politiques gouvernementales de la transition écologique est une aberration. Il faut redonner du sens et des moyens à tous les outils prospectifs et de programmation qui sont à la main des collectivités. Et il faut à cet effet intégrer la transition écologique dans les politiques qui contractualisation avec l’État et proposer des écoconditionnalités partagées et réellement incitatives. À cet égard, le fonds vert, dont nous saluons le maintien dans le projet de loi de finances, manque de transparence et d’articulation avec les politiques publiques territoriales. Il est indispensable qu’une partie des moyens ainsi mobilisés soit affectée à la promotion de stratégies territoriales partagées. Cela permettrait d’éviter le risque de saupoudrage des financements tout en assurant une optimisation de la consommation des crédits. de vue, il faut saluer l’initiative des contrats de relance et de transition écologique (CRTE), qui a été dans l’ensemble plutôt bien accueillie par les collectivités. Une nouvelle génération de CRTE est en préparation. Les attentes sont grandes, car, en particulier, les collectivités ont besoin de visibilité pour engager des investissements. Ces nouveaux CRTE garantiront ils une vision consolidée sur la durée des actions financées par l’État ? Ils devront en effet être bien davantage qu’un programme récapitulant les financements de droit commun des différents ministères ; on en revient aux objectifs et à la conditionnalité. veut avoir davantage de recettes et transformer notre modèle, le principe du pollueur payeur doit être mieux appliqué en France. Cela permettrait de lever les moyens financiers nécessaires à la transition environnementale. De tels montants doivent être largement affectés aux territoires pour leur permettre de piloter les transformations nécessaires, en matière de production comme de mobilités, d’agriculture comme d’aménagement des espaces. Je pense ici aux formidables outils que sont les paiements pour services environnementaux (PSE) et les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui doivent être consolidés auprès des collectivités.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays a traversé récemment des épisodes climatiques extrêmes par lesquels se manifestent plus que jamais

Cet engagement est fondamental pour préparer un avenir habitable non seulement pour les générations futures, mais pour nous mêmes et pour nos enfants. La bonne nouvelle, c’est que nous avons fait la moitié du chemin. La moins bonne, c’est qu’il nous reste sept ans pour faire ce que nous venons de faire en trente trois ans. Pour atteindre l’objectif, pour assumer ce rythme inédit, nous avons un plan. Le secrétariat général à la planification écologique et mon ministère ont travaillé pendant un an à identifier tous les leviers qui nous permettront, secteur par secteur, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre avec la bonne intensité. Cet exercice unique au monde, nous l’avons fait. Ce cadre national, nous l’avons. Désormais, nous devons passer aux travaux pratiques. C’est cela, la déclinaison territoriale de la planification écologique : comment faire pour que les objectifs que nous nous sommes donnés nationalement, et sur lesquels la France s’est engagée, soient effectivement mis en œuvre dans les territoires, par les entreprises, par les Français et, bien entendu, par nos collectivités territoriales ? La Première ministre m’a confié cette responsabilité et je mène, avec ses services, une démarche qui repose sur deux piliers : la mobilisation des citoyens et l’association étroite des collectivités territoriales. La mobilisation des citoyens passe par le tour de France que je mène au plus près des réalités locales. Cet exercice de débat et de pédagogie m’a déjà mené dans sept régions à la rencontre de près de 3 000 Français.

Le tour de France, c’est parler de l’avenir des Français avec eux. C’est leur tenir un discours de vérité et d’humilité, leur dire que chacun de nous a une part de l’effort à faire et une part de la solution entre ses mains.

en affirmant qu’elles sont en première ligne de la transition écologique. J’aime même dire que les maires, réunis en ce moment à Paris, sont les hussards verts de la République. Ils ont un rôle essentiel à jouer,

sont un maillon essentiel de ce que nous sommes en train de mettre en place. Et cela vaut pour tous les échelons, de la région à la commune. Pour embarquer les collectivités dans cette dynamique de planification, nous avons lancé les COP régionales copilotées par les présidents de conseil régional et par les préfets de région. Qu’est ce qu’une COP ? C’est une enceinte de coordination et de travail qui permet aux acteurs régionaux, collectivités, monde économique, monde associatif,

la semaine dernière dans le Grand Est et en Guadeloupe, je veux saluer la dynamique au sein des collectivités territoriales engagées dans ce processus. Évidemment, en tant que parlementaires, vous y serez associés étroitement pendant toute la durée des travaux, qui se dérouleront jusqu’à l’été prochain. Dans les régions non plus, nous ne partons pas d’une page blanche.

poursuivra l’ambition de fédérer les acteurs de la région autour de trajectoires et d’actions communes jusqu’au dernier kilomètre de l’action publique. La territorialisation de la planification écologique doit permettre à toutes les collectivités de s’approprier les objectifs nationaux et de les traduire en projets concrets. Ce dernier kilomètre de la planification nous impose de revoir la manière dont l’État agit avec les territoires. Il nous impose de repenser en même temps les trois dimensions traditionnelles de l’action publique que sont le diagnostic, le portage de projet et l’ingénierie territoriale. le diagnostic, sans lequel rien n’est possible. Aujourd’hui, nous faisons le constat d’un besoin de simplification pour que les collectivités puissent disposer de données et d’indicateurs de transition écologique uniformisés et pertinents. Nous allons outiller les élus et les agents territoriaux en mettant à leur disposition un socle commun d’indicateurs territoriaux facilitant le pilotage de la transition de leur territoire. C’est une dimension clé. Cet outil est déjà disponible. Après la phase de diagnostic, il y a les projets à accompagner. Nous avons une philosophie : pour que le partenariat État collectivités fonctionne en matière de planification écologique, nous devons donner de la visibilité pluriannuelle et adapter

la pluriannualité des financements dans le cadre du recensement des projets participant à la transition écologique. Ne refaisons pas un tour de piste pour savoir quels sont les engagements déjà pris par les collectivités. Assurons nous juste que les « tuyaux » des projets arrivent bien en face des « tuyaux » destinés aux financements. D’autre part, nous allons mieux poursuivre et articuler entre eux l’ensemble des programmes publics de soutien aux collectivités qui permettent de dynamiser les territoires : Action cœur de ville, Petites Villes de demain, Villages d’avenir, Territoires d’industrie. L’ingénierie est une

pour concrétiser un nouvel engagement de cohérence, de coordination et de simplification de l’ingénierie territoriale, souhaité notamment au Sénat à l’occasion d’un rapport sur l’agenciarisation. Enfin, et je terminerai par ce qui est le préalable de toutes nos actions : pour agir, il faut comprendre,

débat interactif. Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l’éventuelle réplique. Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente. Le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à une réplique pendant une minute

le fonds vert aide nos collectivités et leurs groupements à s’engager pleinement dans la transition écologique. Toutes les communes, y compris rurales, peuvent prétendre à ces crédits, et nous nous en réjouissons. Ce fonds est un succès, salué par les élus. Pourtant, certains retours de terrain alertent encore quant à la difficulté d’accès aux subventions. Les démarches restent longues et complexes, surtout pour les collectivités qui sont peu dotées en ingénierie. Prenons un exemple très concret, tiré de mon département, la Marne, et lié à l’éclairage public, sujet qui représente près du quart des dossiers du fonds verts, d’après les chiffres publiés par votre ministère en juin dernier. Pour déposer un dossier visant à rénover son parc d’éclairage public, une commune doit fournir une série d’indicateurs. Je pense en particulier à la puissance totale économisée, à la réduction de la densité surfacique moyenne de flux lumineux installé sur la surface du projet ou encore à la surface de trame noire créée par le projet. des éléments parfois compliqués à obtenir, surtout pour certaines petites communes qui s’appuient sur un réseau d’éclairage public vétuste. De plus, certains élus s’étonnent du fait que les critères du fonds vert outrepassent les normes. Si nous gardons l’exemple de l’éclairage public, la température de couleur maximale demandée pour le fonds est de 2 700 alors que la réglementation impose au maximum 3 000 kelvins. Notre rôle est de continuer à bâtir collectivement un environnement propice à l’adaptation de nos collectivités territoriales au changement climatique. Dès lors, pouvez vous énoncer avec précision vos ambitions pour simplifier les candidatures au fonds vert, afin de permettre à toutes les collectivités de soumettre leurs projets dans les meilleures conditions ? La parole est à M. le ministre.

est que nous avons refusé les appels à projets et les appels à manifestation d’intérêt, afin que le dispositif soit souple. Corollaire de cette souplesse, cela a donné lieu parfois à des souplesses préfectorales qui se sont traduites par des rigidités…

C’est aux communes qu’il revient de définir, après concertation avec leurs administrés, les zones dans lesquelles elles souhaitent implanter prioritairement des projets d’énergies renouvelables. Depuis le 1 juillet 2023, et jusqu’à la fin de l’année 2023, les élus locaux sont donc invités à faire des propositions de zones d’accélération. Il y a un mois, ma collègue Annick Jacquemet interrogeait le Gouvernement sur la publication de décrets visant à mettre en œuvre des ZAER. La ministre de la transition énergétique nous avait alors informés que la définition de ces zones ne requérait pas de décrets. Pourtant, le dispositif manque singulièrement de clarté. Les communes doivent déterminer leurs zones d’accélération avant le 31 décembre 2023. Mais nous avons aussi appris que, passé cette échéance, il restera possible pour les communes de communiquer des zones d’accélération à l’État. Certaines sont actuellement sollicitées avec insistance par leur préfet pour présenter leur carte d’accélération. Que se passera t il en cas de carence de zones ? En particulier, monsieur le ministre, pouvez vous nous confirmer qu’aucun régime de sanction n’est prévu dans le cas où les communes ne désigneraient pas de ZAER ? Dans ce cas, est il par ailleurs prévu que l’État prenne le relais ? Si oui, de quelle manière ? En concertation avec les communes ou unilatéralement ? Nous avons besoin d’éclaircissements. La parole est à M. le ministre. Monsieur le sénateur Pillefer, je suis à la fois ému et touché par votre question, qui concerne plus particulièrement le portefeuille de ma collègue Agnès Pannier Runacher, mais je me ferai un immense plaisir de vous apporter quelques éclairages sur les énergies renouvelables. Vous le savez, nous mettons en nous mettons en France en moyenne deux fois plus de temps que nos voisins allemands pour faire aboutir des projets d’énergie renouvelable. C’est vrai pour le photovoltaïque, pour l’éolien et aussi pour l’éolien offshore. Une loi relative à l’accélération de la production

M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, il faut le saluer, avec votre planification écologique, l’État amorce un virage réel en matière de transition. Ça va un peu plus loin et ça va un peu plus fort : tant mieux ! Néanmoins, le décalage entre l’immensité des besoins et les moyens déployés est réel : 7 milliards en 2024, et encore en recyclant des crédits là où il en faudrait trois fois plus. Le challenge est donc réel. Ce sera l’objet de nos débats lors de En matière de transition écologique, il n’y a pas que l’enjeu stratégie bas carbone. Or, dans vos COP, il n’y a que six mois pour coopérer et deux mois seulement pour construire dans chaque région des diagnostics partagés, qui s’adressent essentiellement – quand on regarde les invités – aux grandes collectivités territoriales. Si nous voulons vraiment associer les collectivités, il faut qu’elles aient les moyens de contribuer. Urgence ne veut pas dire précipitation. Je viens d’entendre votre réponse sur les constructions de diagnostics partagés dans ces COP., si j’ai bien compris votre

quelle est l’articulation avec la feuille de route nationale ? Comment atteindra t on les objectifs qui ont été présentés en septembre ?

projets et ses travaux vous passionnent, je ne peux que vous en faire la publicité et vous inviter à les regarder. Très concrètement, la dotation pour la valorisation des aménités rurales décidée dans le cadre de ce budget, monsieur le commissaire aux finances, aura pour vocation d’accompagner les 88 % du territoire occupé par la ruralité.

puits de carbone, les espaces ruraux représentent d’importants potentiels écologiques sur 88 % de la surface de notre pays. Les collectivités locales, qui sont sans nul doute des rouages essentiels de la transition écologique, sont en première ligne pour faire face aux catastrophes naturelles et aux effets du dérèglement climatique. Nombre d’entre elles sont engagées de longue date dans l’Agenda 21, les plans climat air énergie territoriaux (PCAET), les projets alimentaires territoriaux (PAT), la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations En 2024, le cadre unique et pluriannuel de politique territoriale prendra à l’échelle des intercommunalités la forme d’une seconde génération de contrats de relance et de transition écologique

que les CRTE étaient « améliorables ». La seconde génération de ces contrats annoncée prendra t elle en compte ces critiques ? Comment comptez vous remédier à ces défauts pour que les CRTE soient des contrats intégrateurs porteurs d’un véritable projet de territoire, avec les moyens financiers et en ingénierie adéquats pour les collectivités

président d’une communauté urbaine dans laquelle la plus petite commune comptait moins de 150 habitants, je puis vous assurer que celle ci n’était pas la moins active pour voir comment, à son échelle et à son niveau, décarboner, modifier ou piétonniser une partie de son espace.

Pour cela, les outils et les moyens donnés aux collectivités doivent être à la hauteur. Je pense par exemple aux plans climat air énergie territoriaux, qui semblent un peu à la peine, alors qu’ils sont déployés à l’échelon intercommunal, ce dernier étant certainement le plus adapté pour la planification écologique, puisqu’il est synonyme de bassin de vie. de coopération intercommunale (EPCI) devant réaliser un PCAET avaient lancé la démarche cet été, seuls 57 % d’entre eux l’avaient déjà réellement adopté. Par ailleurs, très peu ont un objectif égal ou supérieur à l’objectif national de neutralité carbone en 2050. Au delà des besoins massifs en investissements et du millefeuille administratif, qui gêne parfois les élus et les agents dans la conduite de leurs projets de transition, il peut exister un manque criant de formation et de sensibilisation des élus aux enjeux environnementaux. La formation, l’accompagnement et l’augmentation des capacités d’ingénierie publique pourraient accélérer la déclinaison territoriale des objectifs nationaux, notamment dans les petites collectivités. Conscients des enjeux et des besoins, les maires ruraux se sont saisis du sujet, à travers un atelier qui a réuni 100 élus volontaires pendant six mois, aboutissant à une position politique de 90 pages, conçue comme une boîte à outils.

D’une part, un tel projet ne semble pas avoir pris l’ampleur espérée. D’autre part, il ne paraît pas concerner les agents publics, qui sont pourtant aussi en première ligne sur ces dossiers. J’aimerais savoir si ces temps de formation pour les maires commencent, selon vous, à porter leurs fruits, et s’ils incluent également les agents des collectivités territoriales. La parole est à M. le ministre.

L’une d’entre elles est l’objet d’une proposition de loi qui sera discutée le 14 décembre prochain. Ce texte sera consacré à la possibilité d’un soutien accru pour les communes les moins bien dotées. Le projet de loi de finances, dont nous commençons l’examen ce jeudi, porte, notamment le fonds vert et une enveloppe spécifique de 500 millions d’euros, forte en la matière. C’est un sujet essentiel pour plus de 10 millions d’élèves, près de 1 million de personnels et pour nos élus. Un récent rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales consacré aux investissements scolaires rappelle que les deux tiers des établissements scolaires ont plus de cinquante ans et que leur rénovation s’impose, à des niveaux divers. Cela passe par un financement accru et par l’accompagnement des élus, notamment ceux des communes les moins peuplées, de moins de 3 500 habitants, en matière d’ingénierie ; il est vrai qu’un projet de rénovation s’apparente parfois à un parcours du combattant ! La planification ne se fera pas sans eux. Dans une circulaire parue le 19 septembre dernier, le Gouvernement a précisé les modalités techniques du programme Villages d’avenir, avec pour objectif un renfort en ingénierie. Concrètement, 100 chefs de projet seront recrutés dans différentes préfectures et sous préfectures, avec la mission d’accompagner les maires à concrétiser leurs idées. À partir de quand les premiers lauréats seront ils annoncés ? Les élus qui n’auront pas été sélectionnés cette fois

favoriser le lien avec la préfecture, faire en sorte de diminuer la paperasse ou les éventuelles difficultés, permettre un accès à l’information dans de bonnes conditions, assurer une veille, vérifier auprès de l’ANCT ou du ministère la disponibilité des financements et l’effectivité de leur mise en œuvre. Quand arrivent Nous avons bon espoir que le projet de loi de finances qui vous est soumis obtiendra une validation globale du Parlement avant le 31 décembre de cette année, ce qui nous permettra de lancer l’ensemble des recrutements

l’emprise urbaine augmente régulièrement : un peu plus de 130 hectares par an, pour un territoire de 2 512 kilomètres carrés. La surface agricole utilisée a diminué de 10 % en dix ans, selon les chiffres de la préfecture. Vous le voyez, il nous faut agir, et chaque année compte pour protéger nos espaces naturels, forestiers et agricoles. Le schéma d’aménagement régional (SAR) de La Réunion doit être finalisé en 2026,

Ce sont de précieuses années que nous perdons, alors qu’il est urgent de protéger nos terres de l’artificialisation des sols, pour préserver tant l’environnement, notamment la biodiversité, que notre sécurité alimentaire. Je rappelle que les terres agricoles sont essentielles pour réduire notre dépendance aux importations de biens alimentaires depuis l’étranger ! Se posent également la question du logement, avec 42 000 demandes de logement social en attente, mais également celle de la pression démographique : La Réunion comptera 1 million d’habitants d’ici à vingt L’exemple réunionnais vaut, très probablement, pour d’autres territoires. Monsieur le ministre, ne faut il pas avancer le calendrier pour la définition du SAR ? Avons nous le temps d’attendre 2026, voire 2027 ou 2028 pour la déclinaison de ces mesures dans les Scot ?

en sorte que des délais supplémentaires soient confiés aux collectivités régionales, en allongeant de neuf mois les temps qui étaient prévus. Je l’assume

l’environnement et l’énergie. L’objectif est de réduire les émissions de CO2 de près de 140 millions de tonnes d’ici à 2030. Le Gouvernement a ainsi prévu de mobiliser 10 milliards d’euros supplémentaires dans le projet de loi de finances pour La stratégie nationale bas carbone mise sur des investissements massifs et rapides des collectivités locales dans de nombreux secteurs, comme les transports collectifs, les infrastructures cyclables ou encore la rénovation des bâtiments publics. Toutefois, les collectivités ne savent pas si elles auront les moyens de faire ce que l’État attend d’elles, sachant que, depuis 2010, les réformes de la fiscalité ont conduit à la réduction, voire à la suppression progressive d’une large partie des recettes. La transformation de la taxe professionnelle, puis la suppression de la taxe d’habitation valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ont réduit la fiscalité directe de 40 milliards d’euros. Seules les taxes foncières permettent aujourd’hui de conserver un pouvoir de taux,

pour les régions, le recul de la consommation aura un impact direct sur les recettes perçues au titre de la TVA. Le système de financement des collectivités est déjà à bout de souffle, monsieur le ministre. lors, comment l’État entend il verser ces 10 milliards d’euros ? Seront ils attribués directement aux régions, aux départements et aux communes ? Enfin, les financements accordés seront ils conditionnés à des résultats de performance énergétique et climatique ?

d’abord vous livrer une de mes convictions profondes au titre de la cohésion des territoires, avant de vous répondre sur le financement.

de conversion à l’agroécologie sur les points de captage. Ce sont autant d’effets de levier, car nous misons sur le principe que 1 euro investi par l’État génère 4 euros investis par les collectivités ; 2,5 fois 4 égalent 10. Il nous reste encore un bout à aller chercher.

pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, il nous faudra produire plus d’énergie renouvelable et décarbonée, avec un énergétique équilibré et résilient, ouvert à plusieurs énergies pas seulement à l’électricité – et plusieurs technologies, tout en nous appuyant sur davantage de sobriété énergétique. Un tel travail implique nécessairement une planification territoriale ancrée dans les réalités du terrain. C’est pourquoi l’ensemble des acteurs publics locaux contribuent aujourd’hui, aux côtés de l’État, à la transition énergétique des territoires. Il est impératif de bien coordonner les actions de chacun, afin d’éviter les risques d’incohérence et de perte d’efficacité des interventions. Cependant, de nombreuses collectivités pâtissent d’un déficit d’ingénierie, d’une insuffisance de moyens et d’expertise dans le domaine de l’énergie. Dans ce cadre, il me semble que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) constituent l’outil territorial pertinent pour accompagner les collectivités, tant dans le cadre de la planification énergétique locale – PCAET, zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR) – que dans la mise en œuvre de leurs projets. En effet, elles sont compétentes sur toute la chaîne de valeurs énergétiques et disposent de moyens et d’expertise en matière énergétique. monsieur le ministre, à l’heure où s’engagent les concertations dans le cadre des COP territoriales et où se dessine le futur cadre réglementaire de la planification énergétique, comment mieux reconnaître le rôle des AODE ? La parole est à M. le ministre.

Je crois à la nécessité de développer les énergies renouvelables. C’est incontournable. Je crois à la nécessité de relance de notre programme nucléaire, parce qu’il n’y a pas de dispositif énergétique qui fonctionne sans énergies pilotables et non intermittentes. Derrière, nous

Les collectivités territoriales, départements, intercommunalités, communes, sont aux premières loges, mais elles n’ont – hélas ! – trop souvent plus les ressources pour faire face aux enjeux.

Nous attendons donc que les investissements importants que doivent réaliser les collectivités, avec un mode de validation à définir, puissent être déconnectés des ratios classiques budgétaires – épargne brute, épargne nette, désendettement –, qui bloquent la possibilité d’accéder aux emprunts nécessaires. Cela pourrait être garanti par les intercommunalités, les départements, la Caisse des dépôts et consignations, voire un fonds dédié par l’État. Si cela est vrai pour le patrimoine existant, c’est encore plus pertinent pour les projets d’aménagement en cours ou à venir voulus par l’État ; je pense en particulier aux opérations d’intérêt national. de l’opération qui concerne le plateau de Saclay. Les enjeux liés au développement des connaissances et des savoirs scientifiques de demain, couplés à ceux du développement durable, devraient faire du projet Paris Saclay un dossier expérimental et exemplaire. Logements, voirie, transports en commun, équipements publics, bâtiments de recherche et d’enseignement supérieur et de développement économique sont autant de constructions qui, au delà des normes environnementales qu’elles doivent respecter, doivent aussi servir d’expérimentations et d’exemples. Or la réalité comptable, trop souvent orchestrée par les musiciens de Bercy, érige les bilans des zones d’aménagement concerté (ZAC) comme des murs qui freinent l’action au quotidien de l’ensemble des acteurs, dont les serviteurs de l’État. Monsieur le ministre, quelles modalités financières d’accompagnement prévoyez prévoyez vous de mettre en place pour que cette action de développement soit réellement durable ? La parole est à M. le ministre.

de la transition écologique. La formulation proposée dans le PLF pour l’investissement dans les communes de plus de 3 500 habitants correspond à la position exprimée de manière majoritaire par le bureau de l’AMF. L’étape d’après, c’est la dette verte.

Ce dispositif est en train de se déployer, et je crois profondément que c’est l’un des moyens de parvenir à lever ces deux types de freins. Enfin, pour vous répondre de manière plus géolocalisée, il se trouve que mon directeur de cabinet

progresser dans la transition écologique est une démarche indispensable pour notre pays. Je pense que nous en sommes tous convaincus dans cet hémicycle. Si la France ne se donne pas les moyens d’accompagner le changement, elle devient tributaire de ses conséquences, sur le plan non seulement environnemental, mais également économique. Nos territoires et les habitants sont en première ligne face au changement climatique. Pourtant, lorsqu’il s’agit de la déclinaison territoriale de la planification écologique, nos collectivités locales se retrouvent souvent reléguées au second plan. Deux exemples l’illustrent à mes yeux. Le premier est la multiplication des implantations d’éoliennes dans la ruralité. Je ne compte plus les maires de Moselle qui se plaignent des impacts catastrophiques de celles ci : nuisances sonores, pollution visuelle, artificialisation des sols, souvent pour un rendement plus que négligeable. Or, par une situation cynique, les élus locaux se retrouvent bien souvent contraints d’accepter leur implantation, les retombées économiques directes pour la commune dépassant largement leur dotation globale de fonctionnement.

Comment le texte originel a t il pu ne pas prendre en compte les plaintes émanant des territoires, alors même que nos élus locaux sont les premiers à s’engager au quotidien et concrètement dans la planification écologique, par des projets innovants et souvent adaptés aux conditions locales

C’est le sens de la disparition des appels à projets et des appels à manifestation d’intérêt ; le fonds vert doit garder de la souplesse. C’est le sens de la décision qui a été prise sur la consigne. C’est le sens des décrets auxquels les parlementaires ont été associés et dont nous avons attendu la validation par l’AMF pour les transmettre au Conseil d’État et pouvoir les publier dans quelques jours.

Monsieur le sénateur Weber, je ne suis pas totalement surpris du champ de votre question. Je sais que votre attachement à la biodiversité et aux parcs naturels régionaux ne date pas de votre récente élection au Sénat. Vous êtes même sans doute l’un des rares exemples de

L’objectif de la planification écologique d’atténuer rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, tout en anticipant les conséquences du dérèglement climatique, est un sujet qui – on le pressent – devra affronter sur le terrain une difficile mobilisation de certains d’entre eux, notamment des plus ruraux.

Alors que la territorialisation de la planification écologique, qui doit être menée au pas de charge, prône le débat et la coopération, ils nous rétorquent déjà que les préfets garderont de toute manière et, une nouvelle fois, la main sur les conditions de sa mise en œuvre. Leurs propos ne visent nullement à remettre en cause la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la biodiversité et les ressources naturelles ou de s’adapter au changement climatique.

Pourquoi alors, nous demandent ils, ajouter ce qui est perçu comme une énième couche et ne fait qu’accentuer chez eux le sentiment d’être contraints ? Alors que la stratégie nationale bas carbone compte sur les investissements massifs et rapides mis en œuvre par les collectivités, celles par les collectivités, celles ci se posent et nous posent légitimement la question des moyens qui leur seront alloués, notamment en termes d’ingénierie, pour faire ce que l’on attend d’elles. Monsieur le ministre, comment comptez vous convaincre et mobiliser ces élus dans la défiance ? La parole

Il faut donc réfléchir aux conséquences de décisions souvent imprégnées de générosité et de volontarisme. Toute demande normative, toute exigence de planification écologique risque malheureusement de pénaliser nos collectivités locales, qui sont suffisamment sous pression.

La question de la consultation est posée. C’est peut être dans ce sens qu’il faut se diriger. J’en veux pour preuve les collectivités qui consultent leurs citoyens à l’occasion de la révision de leur PLU ou de la mise en place du plan climat. en place du plan climat. Aidons les à le faire et donnons leur une assistance ! Nous avons besoin d’une écologie associant les territoires et les citoyens, non d’une écologie de la norme et de la punition qui ne débouche que sur de nouvelles contraintes

présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au mois de septembre dernier, une circulaire de Mme la Première ministre a précisé les modalités de la déclinaison territoriale de la planification écologique souhaitée par le Président de la République. prévoit l’organisation de COP régionales associant les exécutifs locaux, coanimées par les présidents des conseils régionaux et les préfets de région, avec pour objectif l’établissement d’ici à l’été 2024 d’une feuille de route régionale pour 2030.

Cela étant, les dépenses des collectivités locales, d’un montant de 275 milliards d’euros chaque année, ne prennent en compte que partiellement les enjeux. Environ 70 milliards d’euros sont consacrés à l’investissement, dont la moitié pour les communes et intercommunalités, avec des aides de l’État à hauteur de 20 %, soit 6 milliards d’euros. La circulaire La circulaire évoque un soutien en ingénierie sans que les contours soient précisés. Or le besoin d’intervention des collectivités pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone est chiffré à 12 milliards d’euros par an. L’accompagnement de l’État sera déterminant. La question du verdissement des dotations d’investissement et de fonctionnement – DETR, DSIL, DGF – se pose donc, en complément du fonds vert. Monsieur le ministre, seriez vous favorable à la mise en œuvre de l’écoconditionnalité des aides de l’État, véritable levier de la transition et de la planification ?

monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie au nom de mon groupe tous les collègues ayant animé ce débat. La transition écologique et énergétique est désormais le cadre d’action des collectivités territoriales et, plus largement, notre horizon commun en matière d’intérêt général.

pour garantir une action globalement efficiente. D’ores et déjà, il est indispensable de s’assurer que les collectivités territoriales auront une capacité financière suffisante, dans la durée, pour mener à terme les projets. Ce point est absolument central. Pour financer leur action en matière de transition écologique, les collectivités devront combiner le recours à l’emprunt à des niveaux – il faut en avoir conscience – inhabituels ; la réorientation de certains de leurs choix d’investissement vers la transition écologique l’augmentation de leurs ressources propres par le biais des politiques tarifaires, de prélèvements sur leurs fonds de roulement ou de ce qu’il reste de fiscalité. En outre, les soutiens financiers de l’État, hypothétiques, seront essentiels pour mobiliser la Nation. Aucun de ces leviers n’est facile à utiliser ; ils devront être combinés. En réalité, la situation nécessitera plus que des ajustements ponctuels. Il ne faut pas se mentir, le mur des investissements liés au climat obligera à reconsidérer la structure de l’équilibre financier issu de la décentralisation. On ne passera On ne passera pas facilement de 55 milliards d’euros d’investissement aujourd’hui à 80 milliards d’euros en 2030. À partir de ce constat, quelles sont les difficultés à traiter ? D’abord, le rapport à l’endettement est très variable suivant le type et la taille des collectivités. La nécessité d’emprunter au delà des niveaux habituels, parce qu’il le faudra, sera pour certaines un frein. Ensuite, les collectivités devront faire des arbitrages entre actions liées au climat et investissements plus classiques. Ce chantier restera difficile tant qu’il n’existera pas, avec l’État, une vision partagée du sujet. Nous considérons que le renforcement des soutiens de l’État aux collectivités est indispensable pour la réussite nationale en matière climatique. La nécessité de redresser les comptes publics n’exonère pas l’État d’aider les collectivités pour réussir la transition climatique. L’évaluation et la revue des politiques publiques spécifiques de l’État devraient permettre de trouver des économies, en même temps que des ressources, tout en améliorant les services publics. L’indexation de la DGF sur l’inflation – non prévue à ce jour – et la pérennisation du fonds vert à 2,5 milliards d’euros par an ne suffiront pas à résoudre l’équation financière de l’action climatique des collectivités locales. Pour bien mesurer les conséquences, les projections indiquent que l’encours de dette des collectivités augmenterait de plus de 77 milliards d’euros en 2030 par rapport à 2022. À système fiscal constant, l’aide de l’État sera d’autant plus décisive que la diminution structurelle des ressources des régions et départements est dès aujourd’hui forte, avec des conséquences sensibles sur les aides futures à l’investissement du bloc communal. Notre système de fiscalité locale est il adapté aux besoins de financement de la transition écologique ? Non.

cela a été évoqué – des facteurs de complexité accrue. C’est d’un accompagnement opérationnel que les collectivités ont besoin : de l’ingénierie, qui demandera des ressources spécifiques non disponibles aujourd’hui, jusqu’à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’évaluation de la performance climatique des projets réalisés. Le dialogue entre l’État et les collectivités doit être réinventé en se basant sur des revues de plans pluriannuels d’investissement (PPI) cohérents avec les possibilités locales de financement et les objectifs retenus retenus en matière de climat. La réussite de la transition écologique du point de vue des collectivités passera par des moyens adaptés et par une refonte du dialogue et de la gestion de projets avec l’État. L’amélioration du « pouvoir de vivre » des plus modestes

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que nous puissions avoir aujourd’hui, pour la deuxième fois, un débat sur la situation des finances publiques locales, en amont de l’examen du projet de loi de finances.

Il faut par ailleurs que nous proposions collectivement des solutions aux difficultés que rencontrent actuellement un certain nombre d’élus. Tout cela ne sera possible qu’à la condition de dépasser certaines postures stériles, comme celle qui consiste, trop souvent, à présenter nos collectivités territoriales comme dispendieuses ou irresponsables. La réalité, c’est que le solde budgétaire des collectivités est chaque année peu ou prou à l’équilibre. Leur dette – vous le savez, monsieur le ministre – ne représente que 8 % de la dette publique.

Malgré ces constats, le Gouvernement fait le choix de demander aux collectivités territoriales un effort très important de baisse de leurs dépenses de fonctionnement, de 0,5 % par an en volume, dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour Je crois pouvoir le dire, notre assemblée est un peu lassée des méthodes d’un État qui demande des efforts aux collectivités, tout en continuant à aggraver son propre déficit, et qui revendique de baisser les impôts, en supprimant en réalité les impôts des autres

Monsieur le ministre, j’espère également que vous ne nous dresserez pas une fois de plus le tableau d’une situation dite « globalement favorable » des collectivités tout en nous assurant que le Gouvernement serait le seul soucieux de venir en aide à celles qui pourraient se trouver dans le besoin.

le mode de financement actuel des départements, qui ne repose plus que sur des dotations et les droits de mutation, n’est plus viable. Nous attendons donc du Gouvernement qu’il se saisisse véritablement de la question.

Les collectivités territoriales ne se résument pas, je vous le dis, à des lignes sur des tableurs ! En assumant la plus grande part de l’investissement public, en assurant les services publics locaux,

Stéphane Sautarel et Hervé Maurey évaluaient à 110 milliards d’euros, sur la période 2024 2030, l’effort budgétaire global qu’il faudrait mobiliser en faveur des transports du quotidien pour respecter nos engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur cette question, suivant l’une des recommandations du rapport, la commission des finances proposera, dans le cadre du projet de loi de finances, la création d’un levier de financement pérenne et puissant en faveur des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), avec l’attribution d’une fraction du produit de la mise aux enchères de quotas carbone. Toujours dans le domaine des transports, nous proposerons aussi l’affectation aux départements et au bloc communal de deux fractions de 50 millions d’euros chacune du produit de la taxe sur les autoroutes que le Gouvernement propose d’instituer. Cette nouvelle ressource pourrait leur permettre de financer l’indispensable remise en état de notre réseau routier, pour laquelle – je tiens à le souligner, monsieur le ministre – les moyens ont cruellement fait défaut ces dernières années.

temps ! J’invite le Gouvernement à remettre sur le métier le travail de refonte de la DGF, pour bâtir un système plus lisible, plus simple et plus juste.

avec vous des finances locales. C’est d’abord pour moi l’occasion de saluer le travail des élus locaux, qui s’engagent au quotidien au service des Français. Le premier message que je veux leur communiquer, c’est qu’ils peuvent compter sur le Gouvernement

La Cour des comptes l’a écrit : à la fin de 2022, la situation financière des collectivités était globalement satisfaisante ; leur épargne brute s’élevait à 43 milliards d’euros, soit 9 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Leur endettement est faible et leurs capacités de remboursement s’améliorent. Et le nombre de communes en difficulté a baissé de 23 % entre 2019 et 2022. Pourtant, je dois le dire, je suis souvent surpris de l’écart entre cette situation, objective, et les propos très alarmistes et sans nuance que j’entends parfois sur les finances locales. Je suis bien conscient de l’hétérogénéité des situations des collectivités, et je n’ignore pas que, pour certains élus, les budgets sont difficiles à boucler. Nous devons mieux rendre compte de ces disparités. Je souhaite donc que le rapport sur les finances locales s’enrichisse d’une analyse de la diversité des situations. Cela nous aidera à construire des constats partagés et à sortir de l’idée que les chiffres sont en trompe l’œil et ne reflètent pas la réalité.

les communes seraient soumises à un « étranglement financier » de la part de l’État. La bonne santé financière en 2022 est d’abord le fruit de la gestion responsable des élus locaux ; vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général. C’est aussi la conséquence d’une politique, constante depuis 2017, visant à soutenir les collectivités territoriales. Nous avons ainsi compensé à l’euro près les réformes de la fiscalité locale, qui ont conduit à confier des ressources dynamiques aux collectivités.

Le Parlement a également décidé en 2016 d’indexer automatiquement les bases locatives sur l’inflation, pour garantir aux élus une progression de leurs recettes. Cela contribue aujourd’hui au dynamisme des recettes des collectivités. J’en viens à la DGF

depuis treize ans ! Nous n’avons jamais laissé les collectivités en difficulté seules face aux crises. Pendant la crise sanitaire, 10 milliards d’euros de soutien ont été accordés aux collectivités. Et l’État a protégé les collectivités de la hausse des prix de l’énergie, la baisse de la fiscalité sur l’électricité, le bouclier tarifaire et l’amortisseur.

25 000 ! L’épargne brute du bloc communal à la fin du mois d’octobre continue de progresser par rapport à la même période en 2022. La situation est en revanche moins bonne pour les départements, qui sont significativement affectés par la baisse des droits de mutation à titre onéreux. Heureusement, sur les dernières années, ces mêmes DMTO avaient très fortement augmenté : ils ont doublé en dix ans, et progressé de 25 % entre 2019 et 2022. Grâce à cela, le fonds de roulement des départements était de 6,8 milliards d’euros

Pour l’avenir, notre trajectoire de finances publiques trace un chemin qui est celui de la baisse progressive du déficit public. L’objectif est de retrouver collectivement un déficit inférieur à 3 % du produit intérieur brut d’ici à 2027, comme nous avions réussi à le faire avant la crise du

C’est pourquoi nous devons inventer une méthode nouvelle ; j’y suis personnellement attaché. Nous pouvons identifier ensemble les économies à réaliser, qui bénéficieront à tous, État et collectivités. Cette méthode doit évidemment associer les collectivités territoriales, ainsi que votre assemblée. Qui mieux que le Sénat pour identifier les leviers de simplification et d’économies ? Qui mieux que le Sénat pour reprendre la réflexion sur les dotations de l’État et, plus largement, sur le financement des collectivités, pour qu’elles disposent de ressources adaptées à leurs besoins tout en ayant une trajectoire de dépenses compatible avec, je le dis, l’indispensable redressement de nos finances publiques ? Nous le savons tous, nous avons collectivement des marges de progression. Je pense au premier plan à la complexité de nos organisations, qui nous coûte cher et complique la vie des élus locaux. Je tiens ici à saluer le travail de la présidente de la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation, Françoise Gatel. 2024, nous avons l’ambition de franchir une première étape de réduction du déficit et de maîtrise des dépenses. Le projet de loi de finances reste, pour autant, très favorable aux collectivités. Tel qu’il a été enrichi par l’Assemblée nationale, il nous permettra de continuer à soutenir les collectivités et de les aider à réaliser les investissements nécessaires pour l’avenir. Ainsi, le fonds vert est pérennisé à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Et le plan France Ruralités prévoit le recrutement de chefs de projets ingénierie dans les territoires ruraux. Nous aurons aussi l’occasion de discuter dans les prochains jours de l’évolution des zones de revitalisation rurale (ZRR), à la lumière des travaux des sénateurs Bernard Delcros, Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau. favorable à une extension du zonage pour couvrir davantage de communes que ce qui est aujourd’hui inscrit dans le texte initial et, par ailleurs, pour rendre les reprises d’entreprises éligibles aux exonérations.

DGF. J’aimerais m’arrêter un instant sur la décorrélation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière. Cette mesure issue de l’Assemblée nationale va dans le sens des nouvelles relations que nous souhaitons bâtir ensemble. Elle était attendue par de nombreux élus. Nous avons de nombreux chantiers à ouvrir pour l’avenir : sur la dotation globale de fonctionnement ; sur la visibilité que nous devons aux collectivités ; sur leurs modalités de financement. Autant de sujets que je sais chers au président Raynal En conclusion, je voudrais insister sur un point. Nous ne gagnons jamais à opposer l’État et les collectivités territoriales. Que ce soit pour redresser les finances publiques ou réussir la transition écologique, une seule méthode fonctionne : le dialogue ! Vous pouvez compter sur ma volonté de faire progresser le débat

Il y a quelques années, la DGF avait baissé durant cinq exercices consécutifs ; elle a ensuite été stabilisée, voire très légèrement augmentée, mais insuffisamment dans le contexte inflationniste. Ce contexte est particulièrement violent pour les collectivités. En effet, elles ne disposent plus de marge de manœuvre pour absorber la hausse des coûts, notamment ceux de l’énergie. Le « filet de sécurité » voté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2022 a permis de pallier l’urgence, ce qui était indispensable. Toutefois, les critères d’éligibilité retenus étaient trop complexes pour que le dispositif soit véritablement efficace. Beaucoup d’élus, faisant face au choc inflationniste, ont cru pouvoir en bénéficier, grâce au versement d’acomptes. Ils s’aperçoivent aujourd’hui que ce n’était pas le cas. pas le cas. Il faut comprendre ces élus locaux. Comment pouvaient ils s’imaginer que l’État leur verserait un acompte sur une somme à laquelle ils n’avaient pas droit ? Pour certaines collectivités – j’en citerai quelques unes, nordistes, chères à mon cœur Crochte, Ghyvelde, Cappelle Brouck, Wemaers Cappel, Saint Pierre Brouck, Zuydcoote, Watten… –, la situation demeure alarmante. Les élus que nous rencontrons nous parlent de perte de confiance. Monsieur le ministre, qu’entend faire le Gouvernement pour rétablir cette précieuse relation avec les élus locaux ?

Monsieur le ministre, contrairement à ce que vous avez indiqué, le mandat municipal en cours est particulièrement rude pour les élus du point de vue financier. Depuis le début de ce mandat, ces derniers ont dû faire face aux conséquences de la crise sanitaire, à une inflation galopante et aux revalorisations à deux reprises du point d’indice. Face à cette situation préoccupante, la réponse de l’État n’a pas été à la hauteur. Les conséquences de la crise du covid 19 ont été très insuffisamment compensées, et l’inflation comme les augmentations du point d’indice ne l’ont été que très marginalement.

qui décide paie ! Cessez de prendre des mesures que les communes doivent financer

qui pose problème : les collectivités sont confrontées à des hausses, de l’inflation, des taux d’intérêt, du point d’indice, à des maintiens relatifs de dotations, même si nous avons entendu qu’il fallait sans doute craindre l’avenir, mais aussi – c’est le plus inquiétant – à un retournement, sans doute durable, du cycle. Vous avez évoqué les DMTO, qui sont en chute libre. Je pense aussi à la taxe intérieure de

vous disiez exactement la même chose en 2017 à propos des bailleurs sociaux, ce qui vous a permis de les ponctionner. On en voit le résultat aujourd’hui : on n’a jamais produit aussi peu de logements sociaux en France, et ce gouvernement porte une responsabilité majeure en la matière. de l’argent à nos communes, à nos collectivités, à nos services publics. Tout le monde le dit, tous les maires le disent, ça craque de partout et le service public local est en souffrance. Personne ne pourra nier la responsabilité du Gouvernement dans ce domaine. Je pense à la baisse constante des dotations de l’État, qui ont perdu 15 milliards d’euros depuis 2012, au fait que les charges réelles de fonctionnement de nos collectivités ont augmenté en 2022 de 5,9 %, quand les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 5,2 %. Tout cela fragilise nos communes, qui sont pourtant des sentinelles de la démocratie. Et à chaque fois que notre pays est en difficulté, à chaque fois que le Président de la République et la majorité se retrouvent confrontés à des problèmes, c’est vers les maires que vous vous tournez. Il y a un certain paradoxe à traiter aussi mal les communes et à s’adresser si souvent aux collectivités quand vous avez besoin de sortir de vos difficultés ! C’est la raison pour laquelle beaucoup de questions sont posées aujourd’hui par les maires, alors même que l’État continue de transférer des compétences aux collectivités sans leur allouer les moyens correspondants. Nous souhaitons donc vous interpeller en ce jour de Congrès des maires de France. Comptez vous donner enfin au service public local les moyens de fonctionner correctement et indexer la DGF sur l’inflation, comme le proposent les parlementaires communistes et les sénateurs de notre groupe ? Bonne question

Bilhac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je rencontre, comme vous, régulièrement les maires de mon département, l’Hérault. Lors de ces réunions, le problème de la sécurité est toujours posé.

aussi disparates. Monsieur le ministre, allez vous accorder les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de tous les Français, sur tout le territoire ? Cette mission régalienne de l’État doit être prise en charge par l’État.

au recrutement et au renforcement des moyens de la police nationale dans tous nos territoires. pour la réplique. La sécurité, c’est l’affaire de l’État ; la tranquillité publique, c’est l’affaire des maires. Il ne faut pas tout mélanger ! La délinquance ou le trafic de drogues ne relèvent pas des compétences des maires

Mme Nadège Havet. Monsieur le ministre, l’article 52 de la loi organique du 1 août 2001 prévoit qu’un rapport portant sur la situation d’ensemble des finances publiques locales soit annexé au projet de loi de finances de l’année.

nous prévoyons d’augmenter encore la dotation du fonds vert, qui doit accompagner les stratégies des collectivités concernant la renaturation, le changement de l’éclairage public ou la rénovation des réseaux d’eau : autant de sujets sur lesquels les collectivités doivent agir, et vite.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les relations entre l’État et les collectivités sont au cœur de notre débat. Si l’État compte de nouveau sur les collectivités pour relever le défi de la transition écologique, il doit tenir ses engagements et accompagner les communes dans la mise en œuvre les politiques qu’il a lui même initiées.

Sa suppression enverrait un signal négatif et menacerait les programmes périscolaires. Certes, le nombre de communes bénéficiant du fonds a diminué. Mais cela ne justifie pas de compromettre les politiques locales. De plus, son maintien ne menace en rien nos finances publiques. Au contraire, ce fonds assure la continuité d’activités enrichissantes dont le rôle pédagogique n’est plus à démontrer pour nos élèves. telle décision, prise, comme souvent, sans consultation des élus locaux, suscite à raison le ressentiment des maires. Elle oublie totalement de prendre en compte les besoins spécifiques des territoires. Monsieur le ministre, supprimer ce fonds serait une erreur. L’État doit continuer à accompagner les communes et garantir la qualité de l’offre périscolaire sans contraindre le budget des collectivités. Je vous remercie par avance de vos éclaircissements sur cette question importante pour nombre de communes. La parole est à M. le ministre

2024 sera compliquée : anticipons, car la suite sera impossible sans réforme de fond. Troisièmement, les départements sont en train de retrouver un effet ciseaux mortifère, du fait de la décorrélation de leurs ressources et de l’exercice de leurs compétences, par ailleurs non pilotables.

leur niveau de service public, mais aussi, par voie de conséquence, leurs investissements. Monsieur le ministre, alors que les collectivités jouent un rôle contracyclique essentiel dans notre pays et qu’elles sont essentielles à la transition écologique, ne prenez pas le risque de casser le moteur territorial de proximité,

Les maires, de bonne foi et encouragés par les services préfectoraux, ont sollicité ces acomptes. Pour autant, aujourd’hui, les communes sont loin d’être sorties de l’ornière, et il est compliqué pour elles de rembourser. Les communes demandent

Au sortir d’une campagne sénatoriale qui nous a vus sillonner nos départements respectifs et rencontrer de très nombreux élus, au moment où s’ouvre le Congrès des maires, on mesure dans ce volumineux rapport de façon palpable le profond décalage existant entre la théorie et la pratique, entre le verbe et la réalité. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, semble t il. Les dynamiques sont historiques, les péréquations veillent sur nous, la redistribution est à son comble. Encore un effort, et la félicité nous gagnera… La réalité est tout autre, monsieur le ministre. La triste réalité, que vous le vouliez ou non, c’est que d’une liberté constitutionnelle, pensée et conçue pour garantir la libre administration des communes, l’autonomie financière est devenue une coquille vide dépourvue de tout effet utile pour nos collectivités. La triste réalité, monsieur le ministre, c’est qu’en vingt ans, le modèle de décentralisation à la française a perdu de sa pertinence face à un double mouvement opéré par l’État, qui a consisté à recentraliser le fonctionnement des collectivités locales tout en accroissant en même temps les charges pesant sur elles. Aujourd’hui, réconcilier le pouvoir central et le pouvoir local apparaîtrait comme une œuvre historique pour notre pays ; je pèse mes mots. C’est même devenu, je le crois sincèrement, un véritable enjeu de démocratie. Y êtes vous prêt, monsieur le ministre ?

Vous me demandez si l’État compensera les pertes de recettes. Je le redis, et c’est l’engagement qui a été pris lors de ce comité interministériel, il n’y aura pas de pertes de recettes.

particulièrement la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la CVAE, qui n’a pas été suffisamment compensée et dont il résulte la perte de plus de 1 milliard d’euros pour les collectivités. Ma question porte donc sur l’autonomie financière des collectivités, un sujet cher aux élus, en particulier aux maires, dont le congrès se déroule cette semaine. Par exemple, pour les communes, le coefficient correcteur, censé censé compenser le transfert de la taxe foncière des départements aux communes, sanctionne les communes rurales, qui en moyenne reversent plus d’argent que les communes les plus urbaines. Cette compensation est difficilement acceptable par les maires. Il est nécessaire de renforcer l’autonomie financière des collectivités, qui a un statut constitutionnel depuis 2003 ; Jean Raymond Hugonet l’a rappelé. En effet, la suppression des impôts territorialisés a accru les mécanismes de transferts financiers de l’État pour les compenser. Ils atteignent désormais la somme colossale de près de 36 milliards d’euros, ce qui interpelle sur la gouvernance des finances publiques locales opérée par l’État. Au total, l’autonomie fiscale des collectivités a été réduite au fur et à mesure des réformes menées par les différents gouvernements depuis 2018, qui ont également causé une perte de lien entre la fiscalité locale et le territoire. Et si le Gouvernement continue sur le chemin de ses dernières réformes, la crainte d’une diminution trop importante de l’autonomie financière des collectivités pourrait aller jusqu’à entraver le principe de leur libre administration. Aussi, monsieur le ministre, qu’envisage le Gouvernement pour permettre une réelle autonomie financière des collectivités ? La parole est à M. le ministre

ont donc amélioré leur situation financière de 6 milliards d’euros. La Cour des comptes insiste notamment sur la situation des départements. Je le redis, ne confondons pas autonomie fiscale et autonomie financière. Je vous suis sur la baisse de l’autonomie fiscale

M. Fabien Genet. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. En guise de compensation, les collectivités territoriales ont vu transférer à leur profit la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prélevée sur leur territoire. Pour assurer l’équilibre à l’euro près, l’État corrige l’écart provoqué par cette compensation en en reversant aux communes sous compensées un montant calculé sur la base d’un coefficient correcteur et prélevé aux communes surcompensées. Dans mon département, la Saône et Loire, 316 communes sur 564 reversent ainsi 33 millions d’euros de fiscalité locale à l’État,

Cette situation est vécue par nombre d’élus locaux comme une perte de lien entre la fiscalité locale et le territoire, mais également comme une forme d’injustice, car ce sont des communes rurales, qui ont le sentiment de payer en faveur des communes urbaines. Bien entendu, il n’est pas question ici de remettre en cause la nécessité impérieuse de compenser les suppressions de recettes locales décidées par le Président de la République ni d’ailleurs de contester la légitimité de la solidarité, voire de la péréquation entre les territoires. Mais vous conviendrez, monsieur le ministre, que nous touchons là à la limite de l’exercice. L’empilement de toutes les réformes de fiscalité locale depuis plus de vingt ans et leurs conséquences, de suppressions en compensations, de transferts en garanties, font que plus personne n’y comprend rien ! Comment comptez vous améliorer les choses ?

Forcées à faire toujours plus avec des moyens de plus en plus contraints, les communes ont de plus en plus de mal à se projeter financièrement avec sérénité.

en l’espèce, pourquoi toujours complexifier les dispositifs d’aides ? En l’espèce, pourquoi ne pas simplement veiller aux engagements initiaux de l’État, en revenant à la compensation intégrale des exonérations de taxes foncières sur les propriétés non bâties ? Ce serait beaucoup plus simple. La parole est à M. le ministre

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons depuis plus d’une heure de la situation des finances publiques locales. C’est heureux, mais il y a bien une situation qui n’est pas florissante : celle des départements.

en 2023, il sera de 58 millions. En 2013, le montant des dotations de l’État était de 182 millions d’euros ; il est aujourd’hui de 129 millions d’euros. Toujours en 2013, les recettes de fiscalité directe étaient de 225 millions d’euros ; elles sont de 48 millions aujourd’hui. Le compte n’y est pas, et un grand nombre de départements est dans la même situation. Les dépenses de fonctionnement ne cessent d’augmenter ; le produit de certains impôts baisse en valeur absolue, particulièrement les DMTO, en raison du retournement du marché de l’immobilier. Dans le même temps, les dépenses liées aux achats de biens et services, la rémunération des agents – sans parler des annonces intempestives –, l’ensemble des prestations sociales et les frais financiers sont poussés à la hausse par des tensions inflationnistes. L’effet de ciseaux – beaucoup en ont parlé – est particulièrement tranchant… Ces dépenses sont structurelles, alors que les recettes sont très volatiles, exogènes et conjoncturelles et qu’elles ne connaissent pas les mêmes dynamiques. Mécaniquement, parce qu’ils ont l’obligation de présenter des budgets en équilibre, la capacité d’investissement des départements se réduit dangereusement, alors que les besoins ne cessent de croître et qu’ils sont des donneurs d’ordre de premier plan. Monsieur le ministre, ce désengagement de l’État et ces transferts de compétences décidés depuis une dizaine d’années et non compensés en totalité rendent la situation intenable.

pour l’année prochaine, comme l’an dernier et comme le prévoit désormais la loi organique. Cet exercice est nécessaire dans un contexte particulièrement incertain pour les collectivités territoriales, comme d’ailleurs pour le budget de l’État. En 2023 et 2024, le ralentissement de l’activité économique devrait limiter la progression globale des recettes des collectivités territoriales, certaines recettes importantes connaissant même une diminution en valeur absolue. Ainsi, selon les prévisions du projet de loi de finances pour 2024, les recettes nettes de TVA, toutes administrations publiques confondues, progresseraient de 4 % en 2023, soit un niveau inférieur à celui de l’inflation. Les recettes de TICPE des régions et des départements pourraient également diminuer sous l’effet de moindres consommations de carburants, dans un contexte de prix toujours élevés des produits pétroliers et de la fin des mesures d’aide de l’État sur le prix des carburants à la pompe. Les recettes de DMTO chuteraient de 20 % à 30 % en 2023. Cette tendance pourrait encore s’aggraver en 2024.

En effet, les collectivités font face en 2023 – et cette tendance se poursuivra, voire s’accentuera en 2024 – à des hausses notables de leurs charges de fonctionnement.

J’évoquerai enfin la hausse des charges des départements confrontés à des dépenses sociales de plus en plus importantes. Le vieillissement de la population expose en particulier les départements à une augmentation durable des dépenses pour l’autonomie, sans compter les dépenses liées au revenu de solidarité active De surcroît, les collectivités vont devoir faire face à des dépenses d’investissement d’ampleur : transition écologique, adaptation et modernisation des transports nécessiteront des financements importants et prolongés. Je rappelle à ce titre que les collectivités détiennent un patrimoine bâti bâti de plus de 225 000 bâtiments pour une surface totale d’environ 280 millions de mètres carrés contre 100 000 bâtiments et 49 millions de mètres carrés pour l’État. Les investissements à réaliser sont donc colossaux Le PLF 2024, comme le précédent, prévoit certaines mesures d’accompagnement comme le fonds vert, le fonds de reconstruction ou encore une nouvelle hausse de la DGF. Pour autant, seront elles suffisantes ? J’en doute, et l’examen du PLF permettra de faire des propositions complémentaires. L’enjeu est de permettre aux collectivités de fournir des services publics de proximité de qualité aux citoyens, de faire face aux changements climatiques, d’accompagner les citoyens les plus fragiles. Est ce nécessaire de rappeler que les transferts financiers de l’État aux collectivités ont pour objectif de permettre à celles ci d’assumer des compétences répondant aux attentes de nos concitoyens ? Est ce nécessaire de rappeler que, pour assumer ces compétences, les collectivités n’ont quasiment plus de ressources fiscales propres ?

de moyen terme et une prévisibilité des ressources pour ne pas décourager l’investissement. Il faut aussi, et ce point est indispensable, mettre en adéquation les ressources des collectivités avec leurs missions et leurs compétences. Le défi est de taille.